à la campagne nationale d'occurrence des composés alkyles perfluorés dans les eaux destinées à la consommation humaine, document publié en mai 2011.

par 2 500 entre 2008 et 2020. En outre, comme le souligne l'Anses dans ses recommandations, il n'existe pas à ce jour de valeurs toxicologiques de référence pour tous les PFAS, ce qui empêche la construction de valeurs sanitaires maximales.

au regard de l'enjeu majeur de santé publique que représentent les PFAS, nous jugeons indispensable d'établir des valeurs guides de ces substances et d'effectuer des contrôles plus réguliers, ce qui passe par leur prise en compte dans le contrôle de qualité des eaux potables. La parole

identifiant la présence des perfluoroalkyles et des polyfluoroalkyles. En effet, ces substances ne font pas partie des paramètres soumis à l'obligation du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine,

PFAS et leur accumulation dans les organismes des personnes contaminées se sont évidemment poursuivies. Pourquoi ? Parce que ces polluants sont très persistants, que ce soit dans l'environnement ou chez les êtres vivants.

Ces amendements tendent à rendre obligatoire la recherche des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées dans les eaux destinées à la consommation humaine. Cette recherche aurait notamment une incidence sur le coût de l'eau facturé au consommateur, dans une proportion qui n'a pas été évaluée à ce stade. Avant de la systématiser,

Nous devons le prendre en considération. Le contrôle de l'eau destinée à la consommation humaine est actuellement encadré par plusieurs articles du code de la santé publique ; ces dispositions transposent une directive européenne de 1998, qui a fixé un cadre précis à cette surveillance. par l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine, nous avons mentionné aux articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-7 et R. 1321-38 du code de la santé publique les paramètres à surveiller tout au long de la chaîne de production et de distribution

on les ignore. Ce sont des poisons très persistants dans l'environnement, très difficiles à traiter et on n'en a qu'une connaissance très partielle. Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement un rapport dans un délai de douze mois.

les solutions à apporter pour procéder à la dépollution. Je le rappelle, ces substances sont largement utilisées dans le secteur industriel, pour des emplois divers et variés : dans l'industrie textile, comme agents imperméabilisants, notamment

triste surnom de « produits chimiques éternels ». Ainsi, les rejets industriels, la pollution des sols et la pollution des nappes phréatiques dus, d'une part, à la production et aux utilisations passées de ces substances et, d'autre part, à la poursuite de leur utilisation, aujourd'hui

Le problème majeur réside dans le fait que ces composés sont difficilement traitables ; par exemple, les procédés habituels de traitement des eaux, comme l'oxydation chimique, la sédimentation, la coagulation, la filtration ou encore l'irradiation aux ultraviolets ne sont pas complètement efficaces. Voilà pourquoi il faut absolument étudier la question

Afin de lutter contre la pollution aux microplastiques, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, ou loi AGEC, a créé l'obligation d'équiper les lave-linge neufs d'un filtre à microfibres plastiques à compter du 1 janvier 2025. Cette obligation a été introduite par voie d'amendement parlementaire, donc sans la moindre évaluation préalable. Le commissaire européen à l'environnement a rappelé en juin dernier que le règlement communautaire relatif aux exigences en matière d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers et aux lave-linge séchants ménagers n'avait pas prévu d'exigences d'écoconception pour les filtres, « étant donné qu'il n'existait pas de solution technique suffisamment au point et commercialement disponible lorsque les exigences d'écoconception ont été examinées ». L'article 8 de ce même règlement prévoit d'ailleurs que la Commission européenne devra réexaminer ces normes à la lumière des progrès technologiques : elle devra, le cas échéant, présenter un projet de proposition de révision du règlement d'ici au 25 décembre 2025. Ce réexamen devra notamment porter sur la faisabilité et sur l'opportunité de nouvelles exigences visant à réduire le taux de microplastiques des eaux évacuées, comme l'installation de filtres.

Il souligne que ces filtres ne sont pas encore au point et détaille les difficultés sous-jacentes : le nettoyage de ces filtres, l'appropriation par le consommateur, l'entretien et le remplacement des filtres usagés. En outre, l'implication des filtres usagés. En outre, l'implication forte du consommateur soulève deux enjeux auxquels aucune réponse n'est apportée à ce jour. En effet, dans le cas où le filtre ne fonctionne plus, deux solutions sont envisageables : premièrement, le consommateur peut mettre en place un système de contournement aboutissant au retrait du filtre pour assurer le fonctionnement normal de sa machine ; deuxièmement, si le filtre est bouché ou s'il a provoqué un dysfonctionnement de la machine, le consommateur ne peut plus utiliser son lave-linge. lui est alors loisible de le réparer- seuls 40 % des particuliers le font aujourd'hui -ou d'en changer, ce qui contribuerait à accélérer le renouvellement des produits, à rebours du but visé par les pouvoirs publics : favoriser la réparation et l'allongement de la durée de vie

avec la loi visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, adoptée en janvier 2021, d'intégrer au patrimoine commun de la Nation « les sons et odeurs qui caractérisent les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins Après l'ajout de ces éléments dans l'énumération des composantes du patrimoine commun de la Nation, on voit mal comment s'opposer à l'inscription de la qualité de l'eau, tout aussi importante, si ce n'est plus. L'avis de la commission

comme patrimoine commun de la Nation. Y sont cités la qualité de l'air, des sites, des paysages, de la biodiversité, ou encore des sons et des odeurs qui caractérise les milieux terrestres et marins. Il était donc légitime que les députés souhaitent combler cette absence dans la liste générale. Quand bien même l'eau fait l'objet d'un livre spécifique du code de l'environnement,

il s'agit bien de qualité de l'eau, et je ne voudrais pas que l'on en fasse un argument qui ne concernerait que les agriculteurs. Nous sommes tous concernés, y compris les collectivités locales, les entreprises, tous ceux qui consomment de l'eau, qui portent donc une responsabilité vis-à-vis de

focus particulier sur la question agricole, car- je vous rejoins sur ce point -les agriculteurs sont en première ligne sur cette question, même s'ils sont loin d'être les seuls. Les différentes mesures

que l'origine humaine d'un milieu aquatique ou humide ne fait pas obstacle à sa protection et à sa bonne gestion ; d'autre part, à exiger de la restauration de la continuité écologique qu'elle veille à ne pas abaisser la ressource locale en eau non plus qu'à détruire des milieux d'intérêt d'origine humaine. Il a été constaté, tant par la recherche scientifique que par les acteurs des territoires, une confusion sur le sens du mot « naturel » trop de gestionnaires de l'eau considèrent aujourd'hui qu'un milieu naturel aquatique ou humide est forcément sauvage et sans humain. Or la nature en France a évolué depuis des millénaires avec les activités humaines : les lacs, les étangs, les plans d'eau, les retenues, les canaux font aussi aussi partie des écosystèmes, bien que la plupart d'entre eux soient issus d'activités humaines passées ou présentes. Ces milieux d'origine humaine rendent de nombreux services écosystémiques. La confusion assimilant « naturel » et « sauvage » a d'ores et déjà conduit à de regrettables décisions dans de nombreux territoires, par exemple à des destructions ou à des assèchements de lacs ou d'étangs. C'est le cas, en particulier, des chantiers de restauration de continuité écologique qui ne réalisent pas d'étude d'impact sérieuse sur l'hydrologie, l'écologie et l'usage des milieux en place. Face au changement climatique, il est nécessaire de garantir la protection de la ressource en eau sur tout le territoire, pour ses usages tant sociaux et économiques que biologiques et écologiques. Aussi les chantiers de continuité écologique doivent-ils s'assurer que le choix d'aménagement d'un ouvrage ne conduise ni à une perte locale en eau de surface ni à une diminution locale du stockage d'eau souterraine,

à M. Pierre Cuypers. De très nombreux scientifiques montrent que les retenues, plans d'eau, lacs, étangs, canaux biefs, apportent des services écosystémiques aujourd'hui indispensables.

des zones humides. La Coordination nationale eau et rivières humaines (Cnerh) a publié récemment une synthèse de plus de cent publications de recherche qui confirme l'existence de ces services. Or ces écosystèmes d'origine humaine, toujours de petite taille, sont mal protégés par le droit, contrairement aux plus grands. Ils sont détruits sans aucune étude d'impact, d'une part, parce que leur utilité écologique est ignorée,

parfois interprétée, à tort, comme un objectif de retour à une « rivière sauvage ». Cet amendement vise donc à enrichir l'article L. 211-1 du code de l'environnement, qui définit l'intérêt général à travers la « gestion équilibrée et durable de l'eau », afin d'étendre expressément la protection de la loi à à ces milieux.

je ne peux que souscrire à la précision selon laquelle la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est d'intérêt général. C'est d'ailleurs ce que dispose l'article L. 210-1 du code de l'environnement : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. » En revanche, l'intérêt de préciser que les sites et zones humides peuvent être d'origine humaine ou naturelle est moins évident le code de l'environnement ne fait pas de distinction selon l'origine anthropique ou non de ces milieux, d'autant qu'il n'est pas toujours aisé de tracer une délimitation nette de cette origine. Enfin, disposer que le rétablissement de la continuité écologique ne peut qu'augmenter, et non diminuer, la ressource en eau disponible

ne fait pas de distinction selon l'origine anthropique ou non de ces milieux. Certains milieux d'origine humaine sont devenus des milieux naturels par leur abandon, d'autres nécessitent au contraire de maintenir une gestion particulière et régulière pour jouer leur rôle positif. Différencier de manière explicite dans la loi les milieux d'origine humaine des autres et lister les écosystèmes aquatiques ou zones humides d'origine humaine ne peut que conduire à l'oubli

Si le Gouvernement ambitionne de porter ce chiffre à 30 % dès 2022, le présent projet de loi ne fait qu'effleurer le sujet des écosystèmes aquatiques d'eau douce. plus un espace est protégé, plus la biodiversité sera restaurée. L'objectif affiché ici est de faciliter la création et l'extension d'aires protégées pour les écosystèmes aquatiques- rivières, lacs, etc. cette connexion participe indéniablement à la nécessaire reconquête de la biodiversité dans ces espaces. Le présent amendement vise donc à favoriser la réussite de nos objectifs nationaux de protection de la biodiversité, notamment en traitant de l'enjeu des aires protégées.

211-1 du code de l'environnement prévoit d'ores et déjà « la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides », il n'est pas utile d'apporter cette précision qui ne ferait que complexifier la rédaction de l'article, sans gain pour la préservation des écosystèmes. L'avis est donc défavorable. Quel est l'avis

Le citoyen est un acteur clé dans la protection de l'environnement. Chacun, à son niveau, a la possibilité, voire le devoir, d'adapter ses comportements afin de s'inscrire dans une démarche respectueuse de notre trésor commun : notre planète. À cet effet, les initiatives individuelles et collectives sont nombreuses. Les opérations de collecte de mégots de cigarettes en milieu urbain ou de nettoyage des littoraux sont devenues choses communes. Toutefois, celles-ci sont loin d'être suffisantes, sachant que, chaque année, les Français jettent environ 81 000 tonnes de déchets sauvages dans la nature.

? Les auteurs de cet amendement proposent, à titre expérimental, que les conseils départementaux organisent, au minimum une fois par mois, des opérations de nettoyage des lieux pouvant faire l'objet de dégradations liées à l'activité humaine.

qui échappent aux réseaux de collecte et de retraitement.

du Gouvernement ? Les rejets de macro-déchets, les rejets d'eaux pluviales et les déversements des réseaux d'assainissement en cas de forte pluie peuvent effectivement être à l'origine de pollutions. C'est pourquoi le Gouvernement a établi une feuille de route « zéro déchet en mer ».

L'intégration d'une orientation visant à la restauration de ces milieux, dans le cadre de la précision du contenu d'une gestion équilibrée et durable des ressources en eau que cet amendement tend à introduire, induit par ailleurs une valorisation économique des services rendus par la nature. Le

dans la mesure où la préservation des zones humides dispose déjà d'au moins trois assises législatives : le 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement vise la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; l'article L. 211-1-1 du code de l'environnement dispose, depuis 2005, « que la préservation et la gestion durable des zones humides [ ...] sont d'intérêt général », », et que les « politiques nationales, régionales et locales d'aménagement des territoires ruraux et l'attribution des aides publiques tiennent compte des difficultés particulières de conservation, d'exploitation et de gestion durable des zones humides et de leur contribution aux politiques de préservation de la diversité biologique [ l'article 19 du présent projet de loi prescrit d'ores et déjà, à l'article L. 210-1 du code de l'environnement « la préservation et, le cas échéant, la restauration des fonctionnalités naturelles des écosystèmes aquatiques [ ...] dont font partie les zones humides Il n'est pas nécessaire de multiplier des dispositions similaires en de multiples endroits du code, au risque d'affaiblir la lisibilité du droit et de créer de possibles contradictions en cas de formulations différentes. J'émets donc un avis défavorable

Ne pas détruire le patrimoine hydraulique que constituent nos moulins est une volonté légitime, d'une part, parce que l'hydroélectricité constitue naturellement une source d'énergie de premier plan pour notre environnement et notre économie, d'autre part, parce que nos moulins font incontestablement partie du patrimoine culturel.

La restauration de la continuité écologique des cours d'eau est essentielle. Le défaut d'une telle restauration se traduit par une perte d'habitat pour les espèces aquatiques, une baisse du taux d'oxygène dans l'eau, ou encore un réchauffement de la température de celle-ci.

et rappeler la ligne de crête, bien identifiée, de notre groupe Union Centriste, nous refusons une continuité écologique qui conduise à la destruction systématique des retenues et des moulins. Nous défendons une continuité écologique apaisée, permettant de valoriser les moulins et de garantir une production hydroélectrique renouvelable, en associant l'ensemble des parties prenantes dans un dialogue le plus constructif possible. d'une mise en oeuvre trop rigide ayant conduit à la destruction de 3 000 à 5 000 retenues d'eau, en particulier des moulins, dans le cadre des programmes d'aide des agences de l'eau, une politique plus apaisée est possible : elle a été défendue dans un excellent rapport de notre collègue Guillaume Chevrollier,

Aussi le présent article, introduit à l'Assemblée nationale par l'adoption de vingt-neuf amendements identiques, exclut-il la destruction des ouvrages hydrauliques, mettant fin à la continuité écologique destructive précédemment mentionnée.

des travaux de l'Assemblée nationale, rédaction qui consacrait un principe de non-destruction des moulins à eau. Elle est soutenue par des acteurs de terrain, parmi lesquels des propriétaires de moulins ou d'étangs, des agriculteurs et des défenseurs du patrimoine.

permettrait d'engager une politique de la continuité écologique plus apaisée, et de réorienter l'action des pouvoirs publics en faveur de la valorisation des ouvrages, dans une perspective de développement durable et conformément au projet de loi initial, qui dispose que la préservation des

Pour apaiser ce débat, il faut replacer les choses dans leur contexte et à leur juste mesure. Pour cela, il est important de préciser que tous les cours d'eau ne sont pas concernés par cette protection, tant s'en faut. De fait, tous les moulins et installations de petite hydroélectricité ne sont potentiellement pas menacés de destruction. Nous sommes favorables à la recherche d'une conciliation entre cet engagement environnemental et le développement de la petite hydroélectricité en France,

de dialogue et de conciliation en cas de conflit, ainsi qu'à garantir la plus grande transparence lorsque des décisions sont prises. Ainsi toute solution de mise en conformité conduisant à la suppression des capacités de production hydroélectriques ou portant atteinte à l'intérêt patrimonial- ce point tient particulièrement à coeur à mes collègues Sylvie Robert et Jean-Pierre Sueur -devra-t-elle être accompagnée d'un argumentaire de l'administration visant à justifier ce choix. En cas de persistance du conflit, une procédure de conciliation sera engagée. Celle-ci sera pilotée par un référent territorial nommé par le préfet du département. En cas d'échec de cette procédure de conciliation, le Comité national de l'eau sera alors mandaté pour présenter des solutions consensuelles afin de trouver une sortie satisfaisante pour l'ensemble des parties.

Le maintien et la restauration de la continuité écologique est un sujet qui a beaucoup occupé notre commission ces derniers mois. Je salue, à ce propos, le travail accompli par Guillaume Chevrollier dans son rapport d'information

sujet de la possible disparition de cet article à l'issue de la commission mixte paritaire. Compte tenu de ces éléments, j'ai décidé de m'en remettre à la sagesse du Sénat sur l'opportunité d'en revenir à la rédaction de nos collègues députés. à l'amendement n° 1418 de Martine Filleul, il a pour objet la mise en oeuvre d'une procédure de conciliation en cas de désaccord entre un propriétaire de moulin et l'administration, concernant l'obligation de restauration de la continuité écologique. Les travaux de notre commission ont montré à quel point des tensions pouvaient exister dans certains territoires au sujet des prescriptions administratives en matière d'aménagement et d'équipement des ouvrages hydrauliques. Le législateur doit se saisir de ces questions, afin d'assurer une continuité écologique apaisée qui préserve non seulement l'environnement et la biodiversité, mais également les moulins à eau à forte valeur patrimoniale.

Je suis pêcheur dans tous les sens du terme. J'ai toujours attrapé des truites, en haut, en bas. J'ai toujours vu des écrevisses en haut et en bas.

quelques années de pratique dans cet hémicycle nous montrent, madame la ministre, qu'il vaut mieux tenir que courir. Nous avons aussi, dans l'Orne, une histoire avec les moulins. Certaines associations sont très actives, notamment

Mme la ministre.

nationale ont été passionnés, mais les amendements n'avaient pas été suffisamment préparés en amont. Après le vote à l'Assemblée nationale, de nombreux députés,

Vous avez dit, en effet, prendre l'engagement qu'il n'y aurait aucun problème lors de la commission mixte paritaire. Je suis confus de devoir rappeler que le Gouvernement ne siège pas dans une commission mixte paritaire. Il n'y a que des parlementaires, madame la ministre.